avant la lecture, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. de décaler au jeudi 4 août, après-midi et, éventuellement, le soir, la lecture, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement rectificative pour 2022. Acte est donné de ces demandes.

à la réduction de cotisations sociales sur les montants payés, ainsi qu'au rehaussement du plafond de défiscalisation de l'impôt sur le revenu du temps de travail supplémentaire et complémentaire effectué par les salariés, jusqu'à 7 500 euros au titre de l'année 2022,

parole est à M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à rendre éligible le temps supplémentaire des cadres soumis au forfait jours à la réduction de cotisations sociales sur les montants payés, ainsi qu'au rehaussement du plafond de défiscalisation de l'impôt sur le revenu du temps de travail supplémentaire et complémentaire effectué par les salariés, jusqu'à 7 500 euros au titre de l'année 2022, soit entre le 1janvier 2022 et le 31 décembre 2022. l'exonération d'impôt et la réduction de cotisations sociales ne concernent, s'agissant des forfaits jours, que les rémunérations versées pour les jours travaillés au-delà de 218 jours, ce qui exclut de fait plusieurs entreprises mieux-disantes. Il serait pertinent mieux-disantes. Il serait pertinent que toutes les entreprises appliquant un accord de branche ou d'entreprise prévoyant un forfait d'un volume annuel de jours travaillés inférieur à 218 jours

Le coût de la vie ne cesse d'augmenter, comme en témoigne l'inflation galopante de ces derniers mois. La possibilité de travailler le dimanche se traduirait pour de nombreux salariés par une augmentation de leur pouvoir d'achat.

Aujourd'hui, les heures supplémentaires effectuées ne sont pas soumises à l'impôt, dans la limite de 5 000 euros par an, plafond relevé à 7 500 euros. Avec cet amendement, vous revenez indirectement sur la majoration des heures supplémentaires le dimanche, qui est de 25 % les huit premières heures et de 50 % les heures suivantes. Ces majorations de salaire compensent le travail effectué le dimanche. Ainsi les salariés qui travaillent le dimanche dans un commerce de détail alimentaire bénéficient-ils d'une majoration minimale d'au moins 30 %. En défiscalisant les majorations du travail le dimanche, vous ne rendez pas du pouvoir d'achat aux Français. Vous incitez financièrement les employeurs à faire travailler les salariés le dimanche. Vous facilitez le chantage au travail le dimanche, au détriment du droit au repos et à la vie familiale. Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes opposés à cet amendement.

pour être rémunéré parce que les salaires, eux, n'augmentent pas. J'entends la nécessité de défiscaliser et de désocialiser en relevant les plafonds. Monsieur le ministre, vous dites comprendre l'intention.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à majorer la prime de pouvoir d'achat des personnes en situation d'insertion depuis quelques années, afin de valoriser leur parcours. L'insertion est le premier pas permettant à de nombreuses personnes de retrouver le chemin de l'emploi. Leur parcours est souvent difficile et semé d'embûches.

il s'imposerait sans passage obligé par la négociation collective avec les organisations syndicales. C'est là une attaque contre la réduction du temps de travail à 35 heures. heures. En monétisant toutes les RTT acquises les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, le dépassement du temps de travail au-delà de quarante heures est susceptible

Au-delà du mépris pour le repos et la santé des travailleurs, ce sont les 35 heures que l'on met à mal. Acter un possible rachat des RTT, c'est enterrer définitivement la barrière symbolique de travail hebdomadaire. C'est une attaque directe contre l'idée même de partage du temps de travail, donc de partage des richesses. Plus grave encore, instaurer un tel rachat, c'est méconnaître la nature

mais leur capacité à négocier des accords salariaux sera entravée. On sait pourtant que le travail doit être payé à sa juste valeur. Il y a pourtant une manière plus juste, socialement acceptable et digne d'accroître le pouvoir d'achat : augmenter les salaires. C'est pourquoi nous nous opposons

Pourquoi restreindre la liberté du salarié s'il exprime une telle demande ? Quel est l'avis du Gouvernement ? Même avis, pour les mêmes raisons.

Merci

Les salariés peuvent être fidélisés s'ils sont en mesure de bien faire un travail qui est important à leurs yeux, mais aussi reconnu

mettent en péril la santé des Français. Croyez-vous vraiment que la mesure que vous êtes en train d'adopter va aider à conserver le personnel soignant dans les hôpitaux ?

Valérie Pécresse l'avait promis dans sa campagne présidentielle, et Mme Lavarde est honnête et franche quand elle assume vouloir la fin des 35 heures. Le patronat le plus rétrograde et la droite libérale n'ont jamais accepté la réduction du temps de travail. Vous considérez que la vie d'un travailleur n'est pas organisée autour de la conciliation entre son besoin de gagner un salaire et sa nécessité d'avoir une vie en dehors du travail. Mme Pécresse l'avait promis ; le gouvernement Macron-Borne est en train de le faire ! Ce qui se passe cette nuit est très grave. Vous

En fait, en acceptant le provisoire, vous avez ouvert la porte du pérenne. C'est votre zone de convergence avec la droite et la majorité sénatoriale. Vous devrez expliquer demain matin

tous ces amendements ne vont pas assez loin. Si l'on revenait au travail à la tâche, il y aurait une parfaite adéquation entre le besoin des salariés de gagner de l'argent et celui qu'ont les entreprises de faire face à la dure concurrence internationale

mais cette appellation dit une chose essentielle à tous les citoyens : que dans la vie d'un homme ou d'une femme, il y a le travail, il y a la culture,

patron. Lorsqu'on refuse de discuter et d'instaurer du dialogue social sur des réformes comme celle-là, c'est, au fond, qu'on s'attaque aux salariés

l'avons bien vu : la baisse du chômage a créé des revenus supplémentaires pour l'État. Et, encore une fois, le Trésor n'a pas budgétisé cette somme.

Le scrutin est ouvert.

n° 385 rectifié. Cet amendement vise à supprimer la disposition qui permet de ne pas comptabiliser dans le contingent légal ou conventionnel les heures supplémentaires lorsque les jours de RTT en résultant ont été monétisés. Il s'agit de ne pas faire sortir les salariés du champ de la protection de la limitation du temps de travail.

routier (GNR) les activités constituant « le prolongement de l'acte de production », au titre desquelles on retrouve la méthanisation agricole, à savoir l'activité de « production et, le cas échéant, [ ...] la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles ». Ces structures de méthanisation agricole, en plus de participer à la valorisation des coproduits de l'agriculture, sont en première ligne de la transition énergétique de nombreux secteurs consommateurs consommateurs de biogaz, en lieu et place de carburants fossiles, au bilan carbone bien plus lourd. Ces structures participent également à l'accroissement de la souveraineté énergétique de la France et à la diversification des revenus des exploitants agricoles. C'est pourquoi cette activité doit continuer de bénéficier de la taxation spécifique à l'activité agricole.

agricole. Le droit européen autorise les États membres à adopter des niveaux de taxation réduits pour les carburants utilisés pour des usages particuliers, dont les usages agricoles et forestiers. Les tractopelles utilisées dans les unités de méthanisation répondent à cette définition. La méthanisation agricole est l'illustration d'un cycle complet de valorisation des produits et sous-produits agricoles. Les matières premières telles que les effluents d'élevage sont enfin valorisables au travers de leur pouvoir méthanogène, pour donner, à l'issue

Le chef d'exploitation doit aujourd'hui utiliser le montant perçu de la déduction pour épargne de précaution dans les dix années qui suivent pour effectuer des dépenses liées à l'activité professionnelle. Mais cette épargne peut aussi prendre la forme de stock à rotation lente.

31 décembre 2022. La DEP est un dispositif fiscal qui permet de faire face à la volatilité des revenus en réduisant la fraction imposable du bénéfice agricole. Le chef d'exploitation doit utiliser le montant perçu de la déduction pour épargne de précaution dans les dix années qui suivent, afin d'effectuer des dépenses liées à son activité professionnelle. La DEP présente également une souplesse très appréciable. En cas de difficulté, l'exploitant a la possibilité d'améliorer la trésorerie de son entreprise, en réintégrant tout ou partie de la DEP. À l'inverse, dans les bonnes années, il déduit la fraction de son bénéfice imposable. Ce dispositif récent a déjà fait la preuve de son utilité. Nous proposons donc de le pérenniser. La parole

notamment des entreprises de scierie, afin de sécuriser leur avenir. Il prévoit une durée de provision, et seulement de provision, de cinq ans maximum, à échéance de laquelle, si aucune mobilisation n'est intervenue en investissement, les montants provisionnés seraient à nouveau fiscalisés. Un tel mécanisme, en permettant une consolidation des fonds propres, doit donner au secteur la possibilité de renforcer son dynamisme industriel, qui dépend essentiellement de moyens financiers, et notamment du financement de programmes d'investissement. Le dispositif existe en Allemagne et en Autriche et concourt, avec d'autres mécanismes de charges réduites, à la forte compétitivité des entreprises de ces pays par rapport à la filière bois française. Quel est l'avis de la commission ? Madame la sénatrice,

Même avis, pour les mêmes raisons.

que la taxe d'habitation sur les résidences principales, qui s'éteindra définitivement en 2023. Pour mémoire, dans la loi de finances pour 2022, les encaissements nets s'élèveraient

sur l'article. Beaucoup de nos collègues souhaitent reporter d'un an la suppression de la contribution à l'audiovisuel public que- tout le monde en convient -cette dernière est obsolète. Au bouleversement des usages en matière de consommation audiovisuelle s'ajoute la diminution de 600 000 unités du nombre de foyers redevables depuis 2015 et l'augmentation de près de 1 million de foyers exonérés sur la même période. Hier, tout le monde pointait le caractère obsolète de la redevance. Comme cela a été rappelé voilà quelques instants, nos collègues André Gattolin et Jean-Pierre Leleux

autorité parfaitement indépendante, qui nomme les dirigeants de l'audiovisuel public ? Dois-je rappeler que le Parlement donne son avis sur les contrats d'objectifs et de moyens conclus entre l'État et les sociétés de l'audiovisuel public, et qu'il auditionne régulièrement leurs dirigeants

encore les garanties d'indépendance. Ce dispositif est protecteur et doit constituer un premier pas vers une réflexion plus large sur l'avenir de l'audiovisuel public dans notre pays. La

À l'Assemblée nationale, d'aucuns, placés à l'extrême droite de l'hémicycle, considèrent qu'il faudrait supprimer l'audiovisuel public. Ce sont les mêmes qui soutiennent le gouvernement hongrois dans sa lutte contre les médias indépendants La question essentielle que nous devons nous poser est celle des missions de l'audiovisuel public, puis de son financement pour lui permettre d'assurer ses missions en toute indépendance. Vous présentez la suppression de la redevance comme une solution technique. Nous avons plutôt le sentiment que vous avez décidé de réformer l'audiovisuel public par le biais de son financement. Autrement dit, vous avez fait le choix de ne pas donner à l'audiovisuel public les moyens de ses politiques pour lui imposer de les revoir en fonction des moyens que vous lui donnerez

Dans le même temps, la réforme de l'audiovisuel public, annoncée en 2019, a finalement été terrassée par le covid-19, d'où l'interruption des programmes ! Une telle absence de réflexion interroge. Nous devons travailler sur une contribution qui était peu dynamique et ne reflétait plus les usages. La solution adoptée à l'Assemblée nationale, soit le financement par la TVA, ne peut être que temporaire. dispose donc de deux ans pour mener à bien une réforme de l'audiovisuel public adaptée aux nouvelles pratiques et au nouveau paysage audiovisuels, tout en rationalisant la dépense publique, donc en l'adossant cette fois à un financement adapté.

sur l'avenir de l'audiovisuel public, ses missions, ses ambitions, ce qui le distingue des médias privés et ce que les Français en attendent. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de m'exprimer pour expliquer que la fin de la redevance représentait un changement de canal de financement, et non une fin de l'indépendance. Je ne reviendrais donc pas sur ces arguments, qui ont été rappelés aujourd'hui.

82 % des Français regardent les programmes de France Télévisions, tous écrans confondus, chaque semaine, ce qui en fait le premier média des Français. Pour autant, de nombreux défis se posent à l'audiovisuel public. Ils ne datent pas d'hier. pas d'hier. Ils sont nombreux, et ils ont été accentués par la révolution numérique de plus en plus rapide. Le premier est l'éloignement des jeunes de l'audiovisuel. Les données de Médiamétrie montrent la chute continue des audiences des jeunes depuis dix ans. Je ne vous détaillerai pas les chiffres, mais c'est un enjeu prioritaire que de rapprocher la jeunesse de l'audiovisuel, notamment, une stratégie numérique forte.

ans. Lumni propose aussi des programmes éducatifs à près de 2 millions de visiteurs chaque mois. Slash cumule 215 millions de vues chez les 18-35 ans, notamment pour la série. Comment aller plus loin ?

Il y a donc urgence à créer les conditions d'une confiance nouvelle entre les Français et l'audiovisuel, en particulier l'audiovisuel public. Le principal enjeu touche à l'information, à sa qualité, à sa fiabilité, à sa vérification, son impartialité. C'est un enjeu crucial pour l'avenir de nos démocraties, d'autant plus dans un contexte de guerre mondiale de l'information, de manipulation, de possible ingérence étrangère. Cette défiance des Français traduit aussi un sentiment d'éloignement, un besoin que les médias soient plus proches de leurs préoccupations, de leur vie locale, de leur quotidien. Ils attendent davantage de proximité dans les sujets traités, dans les programmes, mais aussi une meilleure représentativité de leurs voix, de leurs histoires, de leurs diversités. L'audiovisuel public a d'ores et déjà pris à bras-le-corps ces enjeux. France 3 et France Bleu ont groupé leurs forces pour lancer un média numérique dédié à la vie locale. Il sera important d'aller plus loin. Nous discuterons ensemble des différentes possibilités pour renforcer encore les synergies entre Radio France et France Télévisions. Il m'importe aussi de dire un mot de la place des territoires outre-mer, qui a été largement renforcée. Oui, nous avons supprimé France Ô,

Il a permis de déployer des programmes ultramarins sur toutes les chaînes de l'audiovisuel public. En 2018, seuls huit programmes ultramarins étaient diffusés en première partie de soirée sur France 2, France 3 ou France 5. Nous en sommes aujourd'hui à plus de quarante premières parties de soirée dédiées à l'outre-mer, cela touche plus de 42 millions de téléspectateurs. Troisième défi, avec la montée en puissance des plateformes américaines en France- Netflix, Amazon, Disney+, bientôt HBO Max HBO Max -, la défense de notre souveraineté culturelle est plus que jamais nécessaire. Or l'audiovisuel public est un puissant financeur de la création française et européenne, avec 500 millions d'euros

Plus globalement, les médias publics sont des acteurs clés de la vie culturelle. Jamais les chaînes privées ne pourront diffuser autant de musique, de concerts, de films de spectacles ou faire la promotion d'autant de livres et d'ouvrages de littérature contemporaine. Comme vous le voyez, les priorités que j'identifie pour l'avenir de l'audiovisuel public sont claires : la jeunesse ; le numérique ; la fiabilité et le pluralisme de l'information ; la proximité et la diversité ; la création et la culture. La mise en oeuvre de cette ambition passera, à n'en pas douter, par l'accélération des coopérations entre les entreprises de l'audiovisuel public. Il me semble qu'il faut clarifier précisément le champ de ces coopérations prioritaires, les bénéfices attendus au regard de nos priorités, avant de trancher la question de l'organisation du secteur. Des synergies par le bas, une, une fusion mettons tout sur la table ; il n'y a aucun sujet tabou. Mais prenons le temps de la concertation. Cette réflexion doit se construire dans le dialogue avec les sociétés de l'audiovisuel public. J'ai aussi entamé une série de consultations avec les groupes de l'audiovisuel public d'autres pays européens pour échanger avec eux sur les enjeux que nous avons en commun.

Pour pouvoir sereinement mener ce travail collectif de réflexion, le Gouvernement souhaite proposer la prolongation d'un an des contrats d'objectifs et de moyens des entreprises de l'audiovisuel public, ce qui nous permettra de prendre le temps nécessaire de bâtir ensemble la feuille de route pour l'audiovisuel public.

notre attachement à l'audiovisuel public, l'enjeu pour la création française, l'indépendance de la presse et des médias. Nous soutenons l'audiovisuel public et nous croyons qu'un audiovisuel public fort est une garantie démocratique dans notre pays. L'autre élément qui ne semble pas faire débat

vous demandez au Parlement de voter très docilement une mesure qui a été décidée par le Président de la République. Cette méthode a été sanctionnée par les électeurs. La verticalité, c'est fini ! Il faut rendre le pouvoir au Parlement, et il faut que nous ayons un débat de fond sur l'audiovisuel public le plus rapidement possible. C'est pour cette raison que notre groupe propose la suppression d'une telle disposition.

aujourd'hui un enjeu majeur pour notre société, face aux concentrations très importantes dans le secteur privé et à la concurrence des plateformes étrangères, que de conforter et de renforcer, en contrepartie, l'audiovisuel public. Madame la ministre, vous chantez la gloire du service public et de ses réalisations, mais vous créez les conditions de son affaiblissement. Souvent, on nous cite l'Europe en exemple.

Mais je crois, pour reprendre une partie des propos de notre collègue Pierre Ouzoulias, que le Parlement se saisit des pouvoirs qui lui sont conférés

l'on supprime la redevance, mais que l'on va se rattraper sur la TVA parce que tous défendraient le même système ... Nous ne défendons pas tous le même système ! Je l'ai souvent rappelé, il y a plus de chaînes de télévision dans n'importe quelle ville de France que de boulangeries.

le secteur du livre et les autres pans de la politique culturelle ne sont pas financés par un modèle de redevance ! Il suffit de pousser la porte d'un théâtre ou de regarder

examiner des mesures sur l'énergie sans discuter de stratégie énergétique, parler de réforme des conditions de travail et du temps de travail sans avoir de débat au fond ou avec les partenaires sociaux, ou encore aborder le devenir de l'audiovisuel sans mener de discussion sur ce que

Je voterai donc évidemment contre ces amendements. Lors d'un dîner de famille, j'ai demandé

Mme la ministre.

davantage de temps pour réfléchir à une nouvelle contribution. Si nous présentons notre proposition aujourd'hui, c'est bien parce parce que le Gouvernement a décidé d'aller extrêmement vite sur cette question. On aurait pu voter les amendements de suppression de l'article 1 et retravailler ensemble à la question plus tard. Nous sommes contraints par un calendrier. Ensuite, monsieur le ministre, si la proposons vous paraît trop dure pour les plus modestes, déposez donc un sous-amendement et relevez le seuil à partir duquel les Français seraient mis à contribution ! Nous sommes tout à fait prêts à l'accepter. si on le veut, tout mélanger quand on parle d'impôts, mais il faut tout de même garder une certaine logique. Lorsque le président de la commission des finances dit ce soir, comme il lui était déjà arrivé de le faire, qu'il s'inquiétait du désarmement fiscal progressif de l'État et de la baisse des ressources publiques, nous devons, me semble-t-il, l'entendre. Avec notre proposition, nous ne créons pas un nouvel impôt. C'est vous qui supprimez une taxe pour augmenter de manière très illusoire le pouvoir d'achat. Nous proposons de remplacer une contribution qui apparaît effectivement aujourd'hui injuste et datée par une nouvelle contribution plus progressive, plus juste et mieux adaptée au financement de l'audiovisuel public, et qui correspond

Les deux impôts des particuliers présentant un rendement suffisant pour remplacer la CAP sont la TVA [ ...] et l'impôt sur le revenu [ ...]. La mission n'a pas recueilli de données permettant de choisir entre ces deux options. » Cela signifie que la mission n'a pas recueilli de données suffisantes permettant d'opter pour la fraction de la TVA.

d'intégrer la demande de la mise en place d'une commission sur le modèle allemand qui aura pour objet d'évaluer le coût des missions de service public public assignées aux opérateurs audiovisuels, de suivre la gestion du dispositif et de tracer une trajectoire pluriannuelle permettant de concilier les enjeux de garantie de financement et l'objectif d'un audiovisuel public indépendant.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.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

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

la solution retenue par l'Assemblée nationale consistant à affecter à l'audiovisuel public, jusqu'à 2025, une fraction de TVA n'est ni pérenne ni stable. Il est donc à craindre que cette option ne permette pas de stabiliser le modèle économique de l'audiovisuel public. Si la suppression de la redevance audiovisuelle se justifie du point de vue du contribuable, elle fait peser une charge inéquitable sur l'ensemble des Français et n'apporte pas de solution fiscale innovante en phase avec les nouveaux modèles économiques des médias numériques. le Gouvernement a fait adopter, au cours du précédent quinquennat, une taxe sur les services numériques qui vise précisément à faire contribuer les nouveaux géants du numérique au financement de nos services publics. C'est pourquoi cet amendement vise, à l'occasion du débat sur le financement de l'audiovisuel public, à doubler le taux de cette taxe, dite Gafam, afin de renforcer ce levier fiscal, qui paraît plus adapté à la réalité des géants du numérique. Quel

de la proposition qui est faite. Deuxièmement, la TSV vise principalement à faire contribuer l'ensemble des acteurs qui tirent profit de la diffusion d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles professionnelles, et qui bénéficient, à ce titre, du soutien du CNC.

de forfait social les abondements de l'employeur aux plans d'épargne entreprise (PEE) et interentreprises (PEI) qui complètent les versements des salariés pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement de l'entreprise ou d'une entreprise du groupe. Cette exonération permet d'inciter les salariés à flécher leur épargne vers le renforcement des fonds propres des entreprises, d'accroître l'actionnariat salarié, qui est un facteur de motivation et de fidélisation des intéressés, et ainsi de favoriser le partage de la valeur dans l'entreprise. Le présent amendement vise dès lors à pérenniser l'exonération temporaire de forfait social prévue par la loi de finances pour 2021.

visent à réduire le champ d'application de la mesure d'amortissement fiscal des fonds commerciaux acquis à la suite de la crise économique provoquée

le législateur ne peut présumer des intentions abusives d'un contribuable alors même que des motifs relatifs à la pérennité et à la transmission de son entreprise ont présidé à ses choix.

prévue par l'administration fiscale, d'exercice d'une activité opérationnelle par la société dont les titres font l'objet d'un pacte Dutreil jusqu'au terme des engagements de conservation. Si une telle condition est souhaitable concernant les sociétés opérationnelles, elle est bien sûr discutable dans le cas d'une société animatrice qui détient des sociétés opérationnelles. L'ajout d'une telle condition s'apparente en effet à une sanction qui limite, de fait, le recours à ce régime dès lors que, si la cesse d'être animatrice, elle entraîne la fin du régime Dutreil, y compris lorsque la détient des sociétés ayant une activité opérationnelle. prévoir que, si la condition d'animation par la n'est plus respectée, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit ne sera acquise qu'au prorata des participations détenues par la dans des sociétés opérationnelles, et non une perte à 100 % du régime.

Il est primordial de faciliter leur organisation matérielle, qui repose sur un parc de véhicules d'intervention et nécessite une grande consommation de carburant. En effet, la consommation de carburant représente un poste de dépenses considérable pour les SDIS, malgré leurs budgets contraints, contraints, largement abondés par les départements. Aussi, il serait nécessaire qu'ils puissent bénéficier d'un tarif réduit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.

de les exonérer de malus pour les SDIS, pourquoi ne pas le faire pour le même type de véhicule relevant d'autres services publics de l'État et des collectivités locales, qui assurent aussi la protection des Français ?

Je remercie notre rapporteur général pour l'avis de sagesse. J'entends vos explications, monsieur le ministre. Toutefois, je maintiens mon amendement, car je pense que le sujet est tout à fait à propos

tout à fait attendu et apprécié par les SDIS et par la protection civile. La parole

de sécurité, de toutes celles et de tous ceux qui luttent contre les incendies. Des discussions budgétaires se sont tenues avec mon collègue Gérald Darmanin dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur. La programmation,

Afin de les soutenir dans leurs missions, et dans la continuité de la lutte contre l'inflation des prix des carburants, cet amendement de Jean-Yves Roux prévoit une « TICPE pompiers », qui consisterait à minorer de 10 % les tarifs de la fraction sur les produits énergétiques autres que le gaz naturel et le charbon perçue en métropole,

Il prévoit, certes, un taux réduit d'accise sur les énergies pour le carburant utilisé par les véhicules des SDIS, mais il n'en fixe pas le niveau. Par ailleurs, cet amendement ne tend pas à modifier le tableau du même code.

la situation des transporteurs. C'est pourquoi il est proposé d'apporter un soutien supplémentaire à ces entreprises, en prévoyant que les aides en question ne sont pas soumises à l'impôt. Quel

dispositif, qui est alimenté par les sociétés concessionnaires d'autoroute sur le fondement de l'article 32 des contrats de concession, il y a automatiquement un droit à compensation susceptible

en prévoyant que les donneurs d'ordres soient soumis à une redevance en fonction de la volumétrie CO2 du transport auquel ils recourent. L'idée est aussi de protéger les transporteurs, pas en leur imposant une taxation, mais en orientant celle-ci vers les donneurs d'ordres, qui commandent aux transporteurs. La mesure consiste à faire remonter le signal prix au niveau de celui qui commande la prestation de transport. Cette taxe est une incitation immédiate à utiliser des solutions de transport plus écoresponsables. Elle n'a pas d'impact direct sur le transporteur.

Il s'agit de faire fonctionner le principe pollueur-payeur pour le transport routier de marchandises, en remontant aux donneurs d'ordres, aux chargeurs, et non pas aux transporteurs, afin de ne pas compromettre les nécessaires capacités d'investissement de ces derniers pour la décarbonation de leurs flottes de camions.

De nombreuses compagnies aériennes effectuent des vols à vide ou très peu remplis, faute de passagers, contraints par la réglementation européenne sur la conservation des créneaux horaires aéroportuaires.

En janvier dernier, la compagnie Lufthansa a averti devoir faire 18 000 vols à vide si la réglementation ne s'assouplissait pas, émettant ainsi 700 000 tonnes de CO2, soit l'empreinte carbone annuelle de 175 000 Français.